Je connais également l'attention que porte le ministre de l'agriculture à cette question et je suis convaincu que, si la réforme est juste, c'est aussi grâce à une meilleure prise en compte des spécificités agricoles. Avant d'entrer dans le détail de la proposition de loi, je souhaiterais replacer cette initiative dans son contexte. L'attention portée aux retraites agricoles ne date évidemment pas de cette législature. Depuis vingt ans, les réformes et les propositions se sont succédé pour améliorer la situation des retraités agricoles et revaloriser les petites pensions.

il y a près de vingt ans, en créant la retraite complémentaire des exploitants agricoles ; il y a bientôt dix ans, en créant la garantie de retraite minimale pour les chefs d'exploitation, dans le cadre de la réforme alors défendue par Marisol Touraine

Pas à pas, nous avons su collectivement préparer et financer ces mesures de revalorisation, qui ont finalement été votées par l'ensemble des groupes parlementaires, avec le soutien de la majorité et du Gouvernement.

Le gain est significatif, puisque les pensions ont augmenté en moyenne d'environ 100 euros par mois, ce dont nous pouvons tous nous féliciter. Cela signifie-t-il pour autant que la totalité du chemin a été parcourue ? Je ne le crois pas. Le régime de retraite des non-salariés agricoles est devenu profondément complexe, additionnant les strates de pension et multipliant les paramètres.

devra définir dans un délai, lui aussi ambitieux, de trois mois les scénarios permettant d'atteindre l'objectif de transformation du système. Nous devrons veiller collectivement à ne pas remettre en cause les droits acquis et à ne pas fragiliser des carrières linéaires qui ne bénéficieraient pas de cette mesure.

possible. Nos agriculteurs et nos agricultrices, plus largement les Français et les Françaises, nous attendent sur cet horizon de justice sociale. Marche après marche, réforme après réforme, nous trouvons ensemble les chemins d'un compromis républicain,

Un an plus tôt, nous avions déjà voté la loi Chassaigne 1, qui relevait de 75 % à 85 % du Smic la garantie de pension des chefs d'exploitation justifiant d'une carrière complète accomplie en cette qualité.

constitue donc la troisième pierre que la Nation doit apporter à l'édifice de sa reconnaissance envers un monde agricole en grande souffrance et pourtant si essentiel à la grandeur de la France. Le mode de calcul des pensions de nos agriculteurs, il faut bien le dire, est particulièrement illisible. À une pension forfaitaire de 312 euros par mois pour une carrière complète s'ajoute une pension proportionnelle calculée dans le cadre d'un système hybride fonctionnant par points, mais intégrant nombre de paramètres des régimes par annuités, notamment en matière d'âge d'ouverture des droits, de durée d'assurance, de surcote et de décote et de revalorisation des pensions. La pension de base des assurés ayant atteint le taux plein est ensuite portée, au travers de la pension majorée de référence (PMR), à un montant minimum de 748 euros par mois, soit le montant du minimum contributif majoré des régimes alignés. Vient ensuite la pension de retraite complémentaire, également exprimée en points. Les seuls chefs d'exploitation justifiant de la durée de cotisation requise pour l'obtention d'une pension à taux plein,

Les polypensionnés, qui représentent plus de 80 % des assurés du régime, perçoivent des pensions généralement supérieures à celles des monopensionnés. Comment cette situation s'explique-t-elle ? Assez logiquement, elle résulte de la faiblesse des revenus professionnels des agriculteurs. Je rappelle à cet égard que près des deux tiers d'entre eux ne parviennent pas à atteindre le niveau du Smic annuel. Leur effort contributif s'en trouve donc nécessairement amenuisé par rapport à celui des salariés ou des artisans et commerçants, dont les taux de cotisation sont supérieurs. Dans ce contexte, il convient de s'interroger sur l'opportunité de maintenir une des spécificités du régime des non-salariés agricoles en matière de calcul des pensions, à savoir son fonctionnement par points, qui fait reposer le montant de la pension sur l'ensemble de la carrière, tandis que celle des ressortissants des régimes alignés, d'un système par annuités, est calculée sur le fondement des seules vingt-cinq meilleures années de la carrière. En effet, il s'agit, avec le régime des professionnels libéraux, dont les affiliés ne connaissent généralement pas les mêmes difficultés financières, du seul régime de base à fonctionner de la sorte. Fort heureusement, l'inspection générale des affaires sociales (Igas) s'est déjà penchée sur le sujet voilà plus de dix ans. Son rapport, bien que devenu en partie obsolète compte tenu, entre autres, des multiples revalorisations des minima de pension intervenues depuis sa publication, nous éclaire suffisamment sur ce scénario. Il ressort de ces travaux que l'instauration d'un régime par annuités favoriserait les retraités les moins modestes au détriment des plus fragiles. En effet, la bascule impliquerait l'abandon du barème d'attribution des points actuellement en vigueur au profit d'un mode de calcul fondé sur l'application d'un taux au revenu annuel moyen des vingt-cinq meilleures années. Or ce barème est particulièrement redistributif et très protecteur pour les assurés situés en bas de l'échelle des revenus. À moins qu'ils ne bénéficient de la PMR, qui leur assure un taux de remplacement supérieur à 50 %, les assurés aux revenus inférieurs à 12 500 euros par an verraient leurs droits diminuer, tandis que les agriculteurs aux revenus plus élevés bénéficieraient d'un taux de remplacement supérieur au taux plein de 50 % appliqué dans les régimes alignés. De plus, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux ne seraient plus en mesure de valider quatre trimestres par an, comme le leur permet leur assiette de cotisation actuelle, si les règles de validation des trimestres des régimes alignés leur étaient appliquées. Il en résulterait une diminution de leur durée de cotisation et, dans certains cas, la perte du bénéfice de la PMR. Ce n'est pas le sens que nous voulons donner à cette réforme. Nous préconisons donc de retenir la solution identifiée par l'Igas comme la mieux à même de limiter le nombre de perdants, à savoir l'application de la règle des vingt-cinq meilleures années, tout en conservant un fonctionnement par points. Concrètement, il s'agirait de calculer la moyenne annuelle des points acquis au cours des vingt-cinq meilleures années et de l'appliquer à chaque année de la carrière, comme si l'assuré avait obtenu ce même nombre de points chaque année du début à la fin de son activité. Sous réserve d'une réactualisation nécessaire des travaux réalisés voilà dix ans, les retraités du régime agricole pourraient voir leur pension augmenter de près de cinquante euros par mois en moyenne. Le coût de la réforme pourrait atteindre jusqu'à 470 millions d'euros à l'horizon 2030, mais sans doute bien moins en réalité du fait des différentes réformes des minima de pension des retraités agricoles menées en 2014, en 2020 et en 2021, qui ont absorbé une partie du coût évalué en 2012. Quoi qu'il en soit, le régime a les moyens d'assumer une telle charge : en maintenant la part de ses ressources, actuellement supportée par la solidarité nationale, son excédent devrait approcher les 800 millions d'euros en 2026. 2026 est précisément l'horizon auquel le texte, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, fixe l'objectif de mise en oeuvre d'un mode de calcul des pensions de retraite des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq meilleures années. De fait, la MSA n'était techniquement pas en mesure de mettre en oeuvre un tel changement avant cette date. Aux termes de la proposition de loi, il reviendrait au Gouvernement de déterminer par décret les paramètres exacts du nouveau mode de calcul des pensions. Il devra, à cet effet, remettre au Parlement, dans un délai de trois mois, un rapport présentant les options possibles et celle qu'il envisage de retenir, tout en indiquant les dispositions législatives et réglementaires qu'il conviendra de modifier pour permettre son application, évaluant ses conséquences sur le montant des cotisations et des pensions et sur l'équilibre financier du régime, et en proposant des mesures de redistribution et de simplification. Il serait opportun, dans ce cadre, de choisir une montée en charge progressive, de façon à éviter de léser les assurés partis à la retraite juste avant l'entrée en vigueur de la réforme. En outre, le rehaussement de l'effort contributif des assurés, notamment des conjoints collaborateurs, aux fins d'assurer la validation de quatre trimestres par an, mais également des exploitants les moins modestes, doit être envisagé. Les organisations syndicales en ont pleinement conscience et se disent prêtes à y réfléchir. Nous souhaitons également que le mode de calcul de la PMR, notamment en ce qui concerne la prise en compte des pensions de réversion, ainsi que le plafond de revenus qui lui est applicable soient alignés sur ceux du minimum contributif, dans une logique d'équité. Nous y serons attentifs. attentifs. Mes chers collègues, le texte qui vous est soumis est-il parfait ? Bien évidemment, non : j'estime qu'il n'encadre pas de façon pleinement satisfaisante le rôle confié au Gouvernement de définir les paramètres exacts de la réforme. En outre, le délai de trois mois prévu pour la réalisation d'un travail d'évaluation et la formulation de propositions aussi complexes est largement insuffisant. J'ajoute qu'il n'est pas optimal de se prononcer sans évaluation récente et précise des effets et du coût d'une réforme de cette ampleur.

sans garantie d'un nouvel examen ni d'une adoption définitive. Pleinement consciente de l'importance symbolique de cette grande marque de soutien national à ces femmes et à ces hommes auxquels nous sommes tous redevables, la commission a donc jugé préférable de sécuriser les avancées acquises de haute lutte et vous invite à adopter la proposition de loi dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Tous les écoliers de France connaissent par coeur le trop célèbre mot de Sully : « le labourage et le pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée. Pour que l'agriculture demeure à jamais la fierté des Français, adressons aujourd'hui à ceux qui nous nourrissent l'hommage de notre gratitude et de notre considération. La parole

Ainsi, en 2021, la pension minimale des agriculteurs est passée de 75 % à 85 % du Smic, ce qui a permis une augmentation de 120 euros net par mois pour une carrière agricole complète. En 2022, comme l'a souligné Mme la rapporteure, une seconde loi a permis d'étendre aux conjoints agricoles le bénéfice de cette mesure. Or 97 % de ces conjoints sont des femmes, dont la pension moyenne était de 600 euros par mois.

pour une part, de garantir un niveau de vie décent. Malheureusement, ce système ne fonctionne plus notamment en raison de la survenance d'aléas climatiques, des variations des cours des produits alimentaires et des crises sectorielles dont souffre l'agriculture.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le sujet des retraites agricoles a toujours été extrêmement sensible et revient, depuis plusieurs années, au coeur de nos débats. En effet, la faiblesse des revenus des agriculteurs retraités, chefs d'exploitation ou conjoints collaborateurs, pour des carrières que nous savons tous particulièrement dures, exigeantes et pénibles, est choquante. À l'heure où la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations dans le milieu agricole sont devenus des enjeux nationaux de tout premier ordre, il n'est plus acceptable que les non-salariés agricoles perçoivent une pension moyenne inférieure de 700 euros par mois à celle de l'ensemble des retraités. Leur pension de retraite est actuellement établie selon un schéma spécifique, somme d'un empilement de pensions qui se sont ajoutées les unes aux autres au fil des évolutions législatives tentant de remédier à cette criante injustice. Comme souvent dans notre pays, le résultat est d'une complexité inégalée et presque inutile, puisque ces retraités ne perçoivent toujours pas des pensions dignes de leur carrière professionnelle.

Cette disposition semble d'autant plus pertinente que les exploitants sont soumis, plus encore que d'autres professionnels, aux aléas de la nature. Elle est logique à condition de ne pénaliser aucun cotisant et donc sous la réserve d'en mesurer les effets en amont. À ces conditions, elle emporte l'adhésion des sénateurs centristes, dont mon collègue Alain Duffourg

elle ne varie pas d'un centime ! Tout cela a engendré une immense confusion chez les retraités de l'agriculture, beaucoup de frustration et un sentiment d'abandon, alors qu'il fallait au contraire redonner de l'attractivité aux carrières

Nous sommes à la croisée des chemins, entre les calculs en points et les calculs en trimestres, pour des travailleurs qui relèvent souvent simultanément de plusieurs régimes et qui se perdent dans ces méandres mathématiques. Nous atteignons les limites du système en constatant que les retraités de l'agriculture ayant obtenu une retraite complète pour pénibilité ou handicap, donc des points supplémentaires liés à leur situation de santé, ne sont pas éligibles aux dispositions de la loi Chassaigne, qui

présente proposition de loi n'est donc que la réparation d'une injustice que la profession dénonce depuis des décennies. À ce titre, elle est essentielle. Alors que le régime général s'applique à l'ensemble des salariés et des indépendants, les agriculteurs non-salariés, c'est-à-dire les chefs d'exploitation, les collaborateurs d'exploitation, leurs conjoints ou les aides familiaux,

comme le souligne le député Julien Dive, rapporteur à l'Assemblée nationale sur cette proposition de loi, que je tiens à remercier. Le régime de retraite des non-salariés agricoles s'est historiquement construit en marge du régime général de la sécurité sociale et il nous faut collectivement réparer ce désavantage. Car oui, il y a puisque ce mode de calcul engendre une différence flagrante d'indemnités : 1 150 euros brut en moyenne pour les non-salariés agricoles contre 1 500 euros brut en moyenne pour l'ensemble des retraités, soit 350 euros d'injustice ! On ne le répétera jamais assez

en vigueur du dispositif a été reportée à 2026 pour permettre à la MSA d'adapter son système d'information. Adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale en décembre dernier, je suis persuadé que ce texte fera également l'unanimité au Sénat. Nous devons envoyer un signal fort de solidarité envers la profession et communiquer enfin sur un point positif. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des sénateurs de mon groupe voteront cette proposition de loi.

Produits laitiers, fruits et légumes, viande, céréales et légumineuses, voilà quelques produits de première nécessité que chaque Français trouve chaque jour sur sa table grâce à nos agriculteurs, qui travaillent dur pour nous procurer la nourriture que nous consommons toute l'année. Ces produits de qualité, nous les devons entre autres au travail de Jacky, éleveur laitier,

Tous ces travailleurs sans relâche, que je connais personnellement, ont nourri les Français bien souvent 365 jours par an, avec des congés quasi inexistants. Le service rendu, vous en conviendrez, mes chers collègues, au-delà de la richesse produite, est inestimable. En sommes-nous suffisamment conscients et reconnaissants ? À l'heure où notre souveraineté alimentaire donne des signes d'inquiétude, où il nous faut encourager ceux qui consacrent leur vie à ce métier fondamental, quel sort notre société réserve-t-elle aux travailleurs de la terre ? Au regard des montants de retraite que je viens de citer, il n'est pas glorieux Certes, le système de retraite des non-salariés agricoles est un montage complexe, fruit de compromis historiques successifs reposant sur des bases de calcul qui ont évolué au cours du temps. Cependant, comment faire perdurer un décompte aussi obsolète ? Comment justifier la prise en compte de l'intégralité de leur carrière, alors qu'ils sont les premiers confrontés à des aléas climatiques et sanitaires, un revenu zéro et à une première année d'installation blanche ? Et cela alors que la majorité des Français bénéficient de la prise en compte des vingt-cinq meilleures années. Mettre fin à cette inégalité de traitement nous honorerait, mes chers collègues. Si le principe de cette réforme ne saurait trouver d'opposants parmi nous, sa mise en oeuvre n'est en revanche pas si simple et requiert prudence, finesse juridique et délais d'évaluation. Prudence, car il convient de bien peser les conséquences de cette réforme pour qu'elle ne puisse en aucun cas se révéler défavorable aux agriculteurs. Finesse juridique, car il s'agit d'une articulation subtile entre la loi, qui détermine l'architecture duale du système de retraite de base des agriculteurs, et le règlement, qui prévoit son mode de calcul et son fonctionnement à points. Délais d'évaluation enfin, car cette réforme mettra fortement à contribution les services de la MSA pour retracer toutes les carrières et nécessitera une analyse rigoureuse des situations ainsi que des conditions exigibles en fonction des différents statuts, afin d'aboutir, je l'espère, à un nouveau mode de calcul pertinent. Voilà l'objet du consensus qui s'est dégagé de la rédaction votée à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une position sage, que nous devons tenir, malgré nos tentations d'améliorer le texte, si nous voulons aider les agriculteurs et mettre fin dans un avenir proche à ce mode de calcul dépassé de leur pension. Ne pouvant juger de l'issue de la future réforme des retraites, il convient d'aller au bout de cette proposition de loi et de tenir notre cap, afin de réparer l'injustice faite depuis trop longtemps aux agriculteurs. Aussi, mes chers collègues, dans un esprit de responsabilité, parce qu'ils nous nourrissent et qu'ils méritent toute notre reconnaissance, je voterai bien évidemment ce texte. La

ont amélioré les petites retraites des agriculteurs puis celles des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux. Cette proposition de loi vise à une meilleure prise en compte de la retraite des agriculteurs. Il s'agit d'une mesure d'équité, d'une reconnaissance méritée,

Mme Raymonde Poncet Monge. Monsieur le ministre, mes chers collègues, dans un contexte de mobilisation inédite contre la réforme des retraites, cette proposition de loi nous rappelle, à l'inverse, les nombreux chantiers menés pour améliorer les régimes, en l'occurrence celui des non-salariés agricoles. Améliorée par les lois Chassaigne, même si des effets de seuil et des situations d'exclusion des dispositifs persistent, la situation générale demeure difficile pour une grande partie des retraités du régime.

Selon le rapport de l'Assemblée nationale, un agriculteur ayant validé l'ensemble de ses droits ne touchait, fin 2020, qu'une retraite de 880 euros par mois, quand un retraité du régime général bénéficiait d'une retraite de 1 810 euros. ces deux systèmes étant difficilement comparables, nous préférons nous référer aux régimes de retraite des indépendants, comme le soulignait très justement l'inspection

et d'un calcul de court terme de réduction de l'assiette de revenus et des cotisations afférentes, tout en subissant la baisse tendancielle des prix du marché ainsi que l'accaparement de la valeur ajoutée par les transformateurs et la grande distribution. Les agriculteurs ainsi vu croître leurs difficultés, leur taux d'endettement atteignant 41 % en 2019, selon le ministère de l'agriculture. Le remboursement d'emprunts représente parfois, comme pour les éleveurs de bovins, la moitié du solde de l'exploitant, ce qui explique en partie la faiblesse des revenus d'un grand nombre d'agriculteurs, étranglés et piégés par ce modèle agricole promu par la filière. S'y ajoutent la multiplication et la gravité des aléas climatiques : selon le Groupe les pertes de récoltes liées aux sécheresses et aux canicules ont triplé ces cinquante dernières années en Europe. La situation ne peut que s'aggraver, d'autant que le modèle n'est

Il est probable que le calcul sur les vingt-cinq meilleures années favorise, de façon très différenciée, les plus hauts revenus par rapport aux paysans qui ont eu une carrière plate et qui ont cotisé au niveau de l'assiette minimale. Pour ceux-là, une augmentation de l'effort contributif

les paramètres et le mode de calcul permettant d'améliorer sensiblement les pensions des non-salariés agricoles aux revenus les plus faibles et aux carrières parfois incomplètes. Notre vote en faveur de cette proposition de loi s'accompagne de cette vigilance, afin que les transformations législatives ou réglementaires qui s'ensuivront profitent à tous et que le système gagne enfin en lisibilité, en justice et en solidarité pour renouer avec l'attractivité des métiers agricoles. La parole Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, le calcul de la retraite des non-salariés agricoles est un sujet qui préoccupe les acteurs de la filière depuis plusieurs mois. Ils nous ont alertés à diverses reprises, avec le sentiment de faire face à une injustice depuis de trop nombreuses années. Selon la MSA, 48 % des actifs agricoles pourront faire valoir leurs droits à la retraite d'ici à dix ans. Face à ce défi démographique sans précédent pour l'agriculture française, il était temps d'apporter une réponse à cette injustice. Créé en 1952, le régime de retraite des non-salariés agricoles s'est historiquement construit en marge du régime général de la sécurité sociale. le seul régime à ne pas avoir été aligné sur le mode de calcul de la moyenne des vingt-cinq années de carrière les plus rémunératrices depuis l'intégration des artisans et des commerçants dans le régime général de la sécurité sociale en 1973. Comment un agriculteur peut-il se satisfaire d'une telle situation ? En 2016, la France comptait 1,3 million d'anciens agriculteurs non-salariés, dont 56 % de femmes, pour une retraite moyenne de 900 euros brut par mois. Alors que la pension moyenne de l'ensemble des retraités s'établissait à 1 430 euros brut mensuels sur cette même période, celle des anciens exploitants agricoles apparaît très nettement insuffisante, loin de la moyenne des retraités. Par ailleurs, le faible montant des retraites agricoles renforce les inégalités territoriales en engendrant davantage de pauvreté dans les espaces ruraux, où un retraité sur quatre était un ancien agriculteur en 2017. Mes chers collègues, vous le savez tous, être chef d'exploitation agricole exige une capacité de travail hors normes, une abnégation sans pareille pour se lever à n'importe quelle heure et une pugnacité remarquable face aux aléas et caprices climatiques.

à l'époque irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. Je me réjouis donc que nous examinions cette proposition de loi, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 1décembre dernier. L'objectif de ce faire converger le régime de retraite des agriculteurs et ceux des salariés et des indépendants au travers du calcul de la pension sur les vingt-cinq années civiles d'assurance les plus avantageuses. Toutefois, pourquoi ne pas prendre en compte les vingt-cinq meilleures années de revenus ? Comme vous l'avez souligné, madame la rapporteure, le système d'information de la MSA conserve l'historique des assiettes de cotisations pendant huit ans au maximum. Or reconstituer le revenu moyen des années antérieures sur la base des points attribués reviendrait à mettre en place une nouvelle injustice. Comme vous l'indiquez dans votre rapport, madame Gruny, trente points sont accordés indistinctement à des assurés dont les revenus diffèrent de plus de 7 000 euros par an. Autrement dit, un revenu de 14 000 euros procurerait autant de points qu'un revenu de 7 000 euros. Par ailleurs, un rapport de l'Igas démontrait déjà, en 2012, que le passage d'un régime par points à un régime par annuités favoriserait les pensions les plus élevées au détriment des plus modestes. Un tel régime ne permettrait donc pas d'apporter une réponse juste et convenable. Dans le cadre d'un système par points, appliquer la règle des vingt-cinq meilleures années reviendrait à identifier les vingt-cinq années d'assurance les plus avantageuses. parvenir ? En calculant le nombre annuel moyen de points obtenus au cours de ces années et en l'appliquant à chaque année de la carrière de l'assuré, dans la limite de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein. En résumé, le montant de la pension correspondra donc au produit d'un nombre total de points, calculé selon une méthode basée sur la valeur du point. Un accord a été trouvé sur une réécriture de l'article 1 et un mode de un mode de calcul qui tienne compte des vingt-cinq années civiles d'assurance les plus avantageuses et non plus des vingt-cinq meilleures années de revenu, avec un alignement sur le régime général à compter du 1 janvier 2026,

340 000 retraités. Il est temps désormais de voter en faveur d'une nouvelle méthode de calcul pour que l'ensemble des salariés non agricoles puissent percevoir une retraite plus juste. Dans le contexte politique actuel, que chacune et chacun connaît, je pense que le vote de notre assemblée enverra un signal plus que positif. Le groupe RDPI votera donc pour

veulent légitimement mettre fin à cette injustice, cette proposition de loi relève cependant d'un exercice paradoxal : l'objectif est limpide et nécessaire, mais les voies à emprunter pour l'atteindre sont tortueuses et susceptibles d'ajouter de la complexité à un régime de retraite déjà peu lisible. Notre collègue Raymonde Poncet Monge a d'ailleurs évoqué, lors de nos travaux, un rapport de l'Igas de 2012 qui illustre le défi que se donne la présente proposition de loi. Ses auteurs y soulignent que « l'on ne peut considérer de façon isolée une règle d'un régime de retraite sans examiner l'ensemble des règles de ce régime : un alignement limité à une règle n'est pas une garantie d'équité et peut, au contraire, être inéquitable si certaines règles sont introduites sans d'autres qui constituent leur contrepartie. Si le régime des non-salariés agricoles doit être réformé, cette réforme ne devrait donc pas porter sur la seule règle du calcul sur les vingt-cinq meilleures années, mais sur la globalité du régime Notre projet de changer la règle de calcul des pensions agricoles porte donc en creux une très grande ambition. Le régime des non-salariés agricoles est en effet une machine complexe, qui a pour caractéristiques, d'une part, de reposer sur un système de points, d'autre part, de se composer d'une retraite de base ainsi que d'une ou de plusieurs retraites complémentaires, à leur tour éventuellement complétées d'une épargne retraite collective ou individuelle. Cette complexité a une histoire.

Il y soulignait toutefois que « le système n'a[vait] été conçu que dans un objectif de protection sociale minimale pour éviter autant que possible le prélèvement sur les revenus agricoles. » À cette époque, le système en question ne comportait « qu'une seule prestation, l'allocation de vieillesse agricole, d'un montant uniforme, et égal à la moitié de l'allocation aux aux vieux travailleurs salariés ». Nous parlons donc d'un régime social agricole en proie, dès ses origines, à une tension entre assurance privée et assurance sociale. Nous travaillons aujourd'hui à résoudre cette tension : les professions agricoles sont des parties prenantes actives et indispensables à l'aménagement de leur régime de retraite, de manière à ce qu'il évolue vers les mêmes principes que le régime général. Malgré l'objectif partagé par les parlementaires et les retraités, actuels et futurs, du monde agricole, beaucoup reste à faire pour que la situation nous semble satisfaisante. Si les lois Chassaigne nous ont permis d'avancer en ce sens, c'est leur acquis que le présent texte veut encore améliorer. L'apport de ces lois est effectivement considérable pour ce qu'elles ont permis d'inscrire coup sur coup dans le marbre. En 2020, la première loi Chassaigne revalorise le complément différentiel de retraite complémentaire des chefs d'exploitation à hauteur de 85 % du Smic net agricole. Elle concerne les anciens chefs d'exploitation ayant une carrière complète. En 2021, la deuxième loi Chassaigne porte revalorisation de 100 euros en moyenne par mois des plus petites retraites agricoles, des retraites des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux.

L'histoire avait certes mal débuté. Dès mai 2018, le Gouvernement refusait de voter l'amendement d'André Chassaigne visant à faire passer la retraite agricole minimale à 85 % du Smic, au prétexte que cela devait être traité dans la réforme globale des retraites. Ce fut le premier des nombreux actes d'obstruction de l'exécutif sur cette réforme.

J'ai moi-même été saisie par un ancien exploitant agricole. Il m'a indiqué ne bénéficier que d'une augmentation très modeste, car le calcul prend en compte ses bonifications pour enfant. Après avoir espéré atteindre une pension de retraite enfin digne, il a acté qu'il ne recevrait pas plus de 940 euros net de pension par mois. Pour lui, la plus-value de la réforme s'est limitée à un gain de 7,44 euros Ces multiples problématiques posées par le régime des retraites agricoles se manifestent aussi pour les polypensionnés. Michaël Zemmour souligne, dans son livre sur la protection sociale, que leur situation « est souvent désavantageuse (parfois fortement) car elle car elle conduit à prendre en compte dans le calcul d'une partie de la retraite- celle du premier régime auquel on a été affilié -des années de début de carrière, relativement mal payées, et qui auraient été exclues du calcul si les personnes avaient passé toute leur carrière dans le même régime Au vu de ces complexités, nous nous inquiétons pour la définition des modalités de calcul des pensions de retraite agricole sur la base des vingt-cinq meilleures années que prévoit la présente proposition de loi. L'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un amendement disposant qu'un rapport serait remis dans un délai de trois mois au Parlement permettra peut-être d'y voir plus clair et de surmonter l'obstacle technique et législatif, même si, comme notre rapporteure l'a souligné, les délais paraissent courts pour un dossier aussi complexe. Ce rapport présentera, par exemple, les envisagés, les dispositions législatives et réglementaires à modifier, les conséquences sur le montant des cotisations et des pensions et sur l'équilibre financier du régime Creusant ce sillon, l'amendement par lequel notre collègue Raymonde Poncet Monge nous propose une amélioration dudit rapport va dans le bon sens. Il s'agit d'y intégrer des critères visant à favoriser la correction d'une partie des défauts du régime des retraites agricoles, mais aussi de parer les effets pervers que pourrait avoir le calcul des retraites

signalait notamment ses potentiels effets anti-redistributifs : les retraités les plus aisés risquaient ainsi de bénéficier de la solidarité des moins bien lotis, lesquels, eux, cotiseraient en vain. Associer un rapport au passage à la méthode de calcul sur la base des vingt-cinq meilleures années est une réponse intéressante pour éviter de tels écueils. Nous voterons cette proposition de loi, en espérant que les travaux complémentaires attendus permettront une application juste. La

Alors que la pension moyenne des Français s'élève à 1 500 euros, les agriculteurs arrivent à peine à 800 euros, soit en dessous du seuil de pauvreté ! Ces derniers

Pour mémoire, le régime de retraite des non-salariés agricoles s'est construit en marge du régime général de la sécurité sociale. Créé en 1952, le régime de base

Cette pension de retraite proportionnelle fonctionne sur un principe d'acquisition de points cotisés, dont le mécanisme diffère selon le statut de l'assuré. Je vous perds ? ... C'est normal Le régime agricole est incompréhensible, en total décalage avec la réalité et d'une grande complexité, qui n'est en rien justifiée par les spécificités du monde agricole. monde agricole. Les agriculteurs sont désormais les derniers à voir leur retraite calculée sur l'intégralité de la carrière. Ce mode de calcul est une double peine

Rappelons que la retraite des indépendants se calcule sur les vingt-cinq meilleures années et celle des fonctionnaires sur leurs six derniers mois d'activité. Les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de repousser la demande légitime des agriculteurs de voir le calcul de leur retraite fondé sur les seules vingt-cinq meilleures années de leur carrière. En 2021, au salon de l'agriculture, le Président de la République estimait impossible de revaloriser ces pensions de retraite. Non, les agriculteurs ne sont pas des actifs de seconde zone ! La première loi Chassaigne prévoyait la revalorisation des pensions de retraite agricole à hauteur de 85 % du Smic agricole, soit 1 045 euros net. La seconde effectuait un pas supplémentaire afin de revaloriser les pensions de retraite des conjoints et aides familiaux- frères, soeurs et enfants -des exploitants agricoles. Aujourd'hui, permettons aux jeunes agriculteurs qui s'installent d'avoir des perspectives meilleures

Cherchons encore l'erreur, quand on sait que cette même injustice induit une différence de 930 euros entre les retraites des agriculteurs et celles des retraités du régime général

La question du renouvellement des générations en agriculture est en effet essentielle. Nos collègues Laurent Duplomb, Pierre Louault et Serge Mérillou, dans leur remarquable rapport d'information sur la compétitivité de la ferme France, dressent un constat terrible sur la lente érosion de notre agriculture. Certes, la balance commerciale est encore excédentaire de 8 milliards d'euros en 2021, mais pour combien de temps ? ... En vingt ans, la France est passée du deuxième au cinquième rang des exportateurs mondiaux de produits agricoles. Nous sommes l'un des seuls grands pays agricoles dont les parts de marché reculent. Plus inquiétant, en trente ans, plus de 57 % des exploitations ont disparu. Les surfaces agricoles utiles se réduisent et les investissements sont en berne, sans compter les difficultés liées à la transmission des terres et des exploitations.

porteurs de sens et d'avenir. Oui, ces métiers demandent des efforts, mais ils sont passionnants et nos agriculteurs font notre alimentation, en nous vendant des produits de très grande qualité.

il arrive malheureusement que certains d'entre eux soient contraints d'interrompre leur carrière et de partir à la retraite plus tôt, du fait d'une inaptitude physique ou d'une incapacité constatée

et hausse des petites retraites des conjoints collaborateurs d'agriculteurs. J'ai d'ailleurs une pensée particulière pour l'ensemble du travail réalisé par notre collègue député André Chassaigne. Toutefois, il faut aussi s'interroger sur le rythme particulièrement lent de ces évolutions. Alors que l'écart du niveau de retraite entre un agriculteur et un retraité du régime général atteint 930 euros pour des carrières complètes, complètes, ce passage à un calcul sur les vingt-cinq meilleures années pour les retraites des non-salariés agricoles est une bonne chose. Mais n'oublions pas pour autant qu'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur ce passage était prêt depuis mars 2012 et qu'il a totalement été laissé de côté

évidemment, comme l'a rappelé ma collègue Monique Lubin, nous soutiendrons ce texte, qui va dans le bon sens. Nous serons vigilants quant à son application, particulièrement en ce qui concerne les potentiels effets pervers d'une telle réforme sur les petits revenus et sur les personnes ne bénéficiant pas des minima

Mme Frédérique Espagnac, sur l'article. La France compte aujourd'hui 1,3 million de retraités anciens non-salariés agricoles, lesquels bénéficient d'une retraite moyenne de 1 150 euros brut, soit environ 800 euros net, montant bien inférieur à la pension moyenne des autres assurés, qui s'élève à 1 500 euros brut environ. Cette proposition de loi a pour ambition de faire cesser l'injuste mode de calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles. Exploitants agricoles, aides familiaux, collaborateurs, voient leur retraite calculée sur la totalité de leur carrière : une situation bien singulière, qui ne concerne qu'eux. Les lois Chassaigne ont été gages de progrès significatifs, avec la garantie d'un niveau minimum de pension de 1 035 euros, soit 85 % du Smic net agricole. Si j'osais, je dirais que c'est le bon sens paysan qui dictait ces mesures ! Ce même bon sens paysan doit nous mener aujourd'hui à aligner le mode de calcul des retraites des non-salariés agricoles sur le régime de base, en prenant en compte les vingt-cinq meilleures années de leur carrière. À l'heure où le débat sur les retraites occupe la totalité de l'espace médiatique, il est un sujet connexe l'on ne peut passer sous silence : les non-salariés agricoles oeuvrant chaque jour pour nourrir nos compatriotes, dont la pénibilité du travail est incontestable, pâtissent de revenus trop bas. Sans une augmentation significative de leurs revenus d'activité, leurs pensions de retraite resteront beaucoup trop faibles.

porte sur les pensions des compagnes d'agriculteurs déjà à la retraite qui, elles, ne peuvent justifier de vingt-cinq années de cotisations ou qui n'ont quasiment pas du tout cotisé. Nous devrons remettre l'ouvrage sur le métier pour ces femmes. Cette réforme est attendue de longue date,

Selon les paramètres et le financement retenus, elle pourrait aboutir à une dégradation de la solidarité du régime au détriment des paysans

isolé ne va pas sans poser de problèmes, comme indiqué dans le rapport de l'Igas, et n'apporte aucune garantie sur son résultat ni sur son impact différencié. Nous devons au monde agricole la certitude que cette réforme ne pénalisera personne et qu'elle permettra de corriger un certain nombre de dysfonctionnements. Je

ce sens, le délai de remise du rapport devrait être porté à six mois, afin de garantir, en plus d'une analyse précise des modifications à conduire, la consultation approfondie de l'ensemble des parties prenantes lors de l'élaboration de cette étude. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement

De plus, bien que la proposition de loi n'encadre pas suffisamment la compétence confiée au Gouvernement pour ce qui concerne la détermination des modalités de son application, le texte précise d'ores et déjà que le Gouvernement devra proposer des mesures permettant de renforcer la redistribution en faveur des plus fragiles au sein du régime de retraite de base des non-salariés agricoles- ce que souhaitent les auteurs de cet amendement. Enfin, dans le cadre du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le Gouvernement propose plusieurs mesures susceptibles d'améliorer la situation des retraités dont

avant la création du régime complémentaire ou son extension à leur catégorie professionnelle, ou encore le relèvement de 39 000 à 100 000 euros du seuil de récupération sur succession des sommes versées au titre de

l'avis de la commission ? Cet amendement vise à assouplir les critères d'éligibilité au complément différentiel de points de retraite complémentaire des non-salariés agricoles en remplaçant la condition de durée d'assurance par une condition de liquidation à taux plein. Dans la mesure où le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 comporte une disposition de même nature, je vous propose, mon cher collègue, d'examiner cette question dans le cadre de la réforme des retraites à venir et d'adopter le présent texte sans modification.